La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour un rappel au règlement. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur l'article 29

vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue. L'ordre du jour appelle l'examen de quatre projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre et de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l'État plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre

Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d'Équateur sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre (projet n° 66, texte

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la principauté d'Andorre relatif à la coopération technique et

sur proposition de M. Jean-Luc Warsmann et de plusieurs membres du groupe UDI, Agir et Indépendants, l'Assemblée nationale a examiné et adopté après modifications, le 7 décembre dernier, la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen, c'est-à-dire du cadre juridique qui permet l'application du règlement européen du 26 juin 2013, dit « règlement Dublin Cette initiative législative est apparue particulièrement opportune aux yeux du Gouvernement, alors que plusieurs décisions de justice ont ont remis en cause la bonne application de ces mécanismes qui permettent d'organiser la répartition des demandes d'asile entre les pays de l'Union européenne.

la France fait face à une forte croissance, avec 100 000 demandes en 2017, soit une augmentation de 17 %, après des hausses de 6 % en 2016 Et c'est sans compter les 85 000 personnes qui ont fait l'objet d'une décision de non-admission à nos frontières. La demande d'asile est d'abord portée par des nationalités dont le besoin de protection n'est pas très élevé, à l'instar de l'Albanie ou des pays d'Afrique francophone, comme la Guinée ou la Côte d'Ivoire. Mais ce sont surtout les flux de rebond, c'est-à-dire les personnes ayant déjà demandé l'asile dans un autre pays européen et venant tenter leur chance dans l'Hexagone, qui alimentent cette hausse continue de la demande. Jusqu'à une période récente, ces flux de rebond étaient très minoritaires : en 2016, ils représentaient seulement 11 % des demandes d'asile. Mais, depuis quelques mois, la donne a changé. En 2017, 36 % des demandes d'asile en France, soit 41 500 demandes, émanaient de personnes relevant de l'application du règlement Dublin. En Île-de-France, dans les Hauts-de-France, cette proportion a même atteint les 75 %. À titre d'illustration, pour la seule année 2017, le nombre de personnes déboutées du droit d'asile en Allemagne s'est élevé à plus de 230 000, ce qui porte à 500 000 le nombre de déboutés en Allemagne au cours des trois dernières années. Or cette tendance devrait se poursuivre au vu du nombre considérable de personnes déboutées du droit d'asile en Europe, mais n'ayant fait l'objet d'aucune procédure d'éloignement. Mesdames, messieurs les sénateurs, cet accroissement important de la demande d'asile a conduit le Gouvernement à développer de manière substantielle nos capacités d'hébergement. Je rappelle à ce titre que les moyens budgétaires affectés à la mission « Immigration, asile et intégration » ont été augmentés de 26 % dans le cadre de la loi de finances pour 2018 ainsi, nous porterons les capacités du dispositif national d'accueil à 88 000 places à l'horizon 2019, ce qui constituera une augmentation de près de 8 000 places en l'espace de trois ans. Malgré ces efforts, notre système d'hébergement demeure au bord de l'embolie. Pouvons-nous laisser perdurer une situation dans laquelle des milliers de personnes, dont la prise en charge relève pourtant d'autres États, viendraient menacer l'équilibre même de tout notre système ? Chacun mesure que tout cela n'est pas viable. La législation européenne doit être respectée. doit être respectée. Afin de remédier à ces difficultés, j'ai, dès ma prise de fonctions, demandé aux préfets d'appliquer strictement le règlement Dublin en procédant au transfert des personnes vers l'État membre responsable du traitement de leur demande d'asile. obtenu de vrais résultats, puisque le nombre de transferts Dublin a doublé par rapport à 2016, ce qui a permis, dans certains territoires, de soulager nos dispositifs d'hébergement et d'asile. Or, depuis quelques mois, ces progrès significatifs, que nous avions obtenus au prix d'une implication forte de l'administration, se trouvent fragilisés par plusieurs décisions juridictionnelles. Le 15 mars 2017, la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, saisie d'une affaire qui ne concernait pas la France, mais la République tchèque, a invité tous les États membres de l'Union à définir dans leur loi nationale les critères objectifs fondant le « risque non négligeable de fuite » d'un étranger en procédure Dublin, et donc la possibilité d'un placement en rétention. Sur le fondement de cet arrêt, la Cour de cassation a souligné, le 27 septembre dernier, que, si notre droit interne définit bien le « risque de fuite », il devait, pour autoriser le placement en rétention des personnes sous procédure Dublin, préciser ce qu'est le « risque non négligeable de fuite Enfin, le 19 juillet 2017, le juge des référés du Conseil d'État a indiqué que le droit français ne permettait pas au préfet de placer en rétention un étranger soumis au règlement Dublin au cours de la phase de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile. L'effet pratique de ces différentes décisions de justice est d'interdire le placement en rétention de personnes relevant de la procédure Dublin. Il convenait donc d'adopter de nouvelles dispositions législatives,

aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement Dublin peut être placé en rétention. Ce placement ne pourra être décidé que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé, uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si l'assignation à résidence ne peut être effectivement appliquée. À cet effet, le texte définit ce qui caractérise un « risque non négligeable de fuite », par exemple le fait pour l'étranger de s'être déjà soustrait, dans un autre État membre, à l'application du règlement Dublin ; d'avoir déjà été débouté de sa demande d'asile de s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ou encore, pour se maintenir sur le territoire français, d'avoir contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage. De manière très opportune, les députés ont souhaité apporter certaines précisions relatives à la définition de ce risque non négligeable de fuite. À titre d'exemple, si le fait pour l'étranger de dissimuler des éléments de son identité peut caractériser le risque de fuite, il a été ajouté que la circonstance tirée de ce que l'étranger ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation. deuxième axe de cette proposition de loi. L'article 1 transpose en droit interne la possibilité ouverte par l'article 28 du règlement Dublin de placer en rétention administrative un étranger pendant la phase de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, ce qui répond à l'avis du Conseil d'État du mois de juillet dernier. permet également d'étendre les critères d'appréciation du risque non négligeable de fuite lorsque le placement en rétention administrative intervient alors que l'étranger était assigné à résidence et qu'il n'a pas respecté les prescriptions de cette dernière. Je tiens à préciser que des garanties complémentaires ont été apportées lors de l'examen par l'Assemblée nationale. Ainsi, un décret devra préciser les modalités de prise en compte de la vulnérabilité des « dublinés » et, le cas échéant, de leurs besoins particuliers. De même, le présent texte indique désormais que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Au-delà de nombreuses améliorations rédactionnelles et de précisions juridiques, votre commission des lois a, pour sa part, souhaité apporter des compléments au texte de cette proposition de loi. Je comprends les préoccupations que ces compléments traduisent, même si certains d'entre eux pourraient soit paraître éloignés de l'objet de la proposition de loi, soit être d'une efficacité relative. Ainsi, votre commission a introduit un nouveau motif caractérisant le risque non négligeable de fuite applicable si l'étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s'il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement. Pour ma part, je suis sensible au réel problème que pointe cette modification, problème qui, du reste, dépasse la seule question des étrangers soumis au règlement Dublin.

Il envisage de faire des propositions visant à rendre applicable à ce délit la peine d'interdiction du territoire français, dans le cadre du projet de loi Asile et immigration, lequel est actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État. autre complément est proposé par votre commission des lois : la réduction du délai de recours juridictionnel de la décision de transfert Dublin. Actuellement, cette décision peut être contestée dans un délai de quinze jours devant le juge administratif. Votre commission des lois a prévu de ramener ce délai à sept jours, au motif que cette proposition est reprise par la Commission européenne dans son projet de refonte du règlement Dublin, lequel est en cours de discussion. Il s'agit évidemment d'une disposition sensible, mais le Gouvernement comprend le souci d'efficacité qui l'anime. a par ailleurs prévu de porter de quatre à six jours la durée de validité des ordonnances prises par les juges des libertés et de la détention autorisant des visites domiciliaires chez les étrangers assignés à résidence. ont pour objet de s'assurer de la présence de l'étranger à son lieu d'assignation à résidence et de le conduire, le cas échéant, à ses rendez-vous administratifs. Le Gouvernement partage, là aussi, le souci d'amélioration de l'efficacité de ce dispositif introduit dans notre droit par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, même si cette proposition n'est pas directement en rapport avec la problématique des étrangers relevant de l'application du règlement Dublin.

étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, en vertu desquelles l'assignation à résidence des étrangers ayant été condamnés à la peine d'interdiction du territoire français, mais dont l'éloignement est impossible, n'était pas limitée dans le temps. Le Gouvernement considère d'un oeil positif cet ajout, qui comble un vide juridique et opérationnel, dans la mesure où la date du 30 juin 2018 approche à grands pas, même si cet article est lui aussi éloigné de l'objet de la présente proposition de loi. loi. Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement relève que, dans leur totalité, les apports voulus par les députés n'ont pas été remis en cause au terme de l'examen du texte par votre commission des lois,

même si je relève que certaines de ces questions seront traitées dans le cadre du projet de loi Asile et immigration. Nous appelons donc la Haute Assemblée à voter cette proposition de loi dans les termes qui sont proposés

pour reprendre l'application du règlement Dublin, afin de retrouver notre capacité à procéder à des transferts d'étrangers vers les États responsables de l'examen de leur demande d'asile. Comme je l'ai dit en commençant, il s'agit là d'une problématique majeure dans le contexte migratoire que je vous ai exposé. Je veux, mesdames, messieurs les sénateurs, vous remercier.

Cette proposition de loi est courte, son objet est limité et son but est très clair. Il s'agit de résoudre un problème ponctuel, mais urgent : l'impossibilité de placer en rétention et de transférer efficacement les étrangers dont la demande d'asile relève d'un autre pays européen, en application du règlement Dublin. Il est vrai que le régime d'asile européen commun repose sur un principe cardinal : un seul État est compétent pour l'examen d'une demande d'asile. Ce principe a été mis en oeuvre par plusieurs textes européens, le dernier en date étant le troisième règlement Dublin, de 2013.

deuxièmement, lutter contre un éventuel, une course à l'État le plus favorable. Pour déterminer l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, huit critères hiérarchisés sont prévus. Ils prennent en compte la situation familiale du demandeur ainsi que son parcours personnel et migratoire. En pratique, deux critères prédominent. Tout d'abord, l'État responsable de la demande d'asile sera généralement celui qui a reçu la première demande d'asile ou celui dans lequel le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière, terrestre, maritime ou aérienne, de l'espace européen Dublin. Concrètement, le système fonctionne principalement à partir des prises d'empreintes digitales des demandeurs, enregistrées dans la base de données EURODAC. Ensuite, le règlement prévoit les modalités de transfert des étrangers « dublinés » vers l'État responsable du traitement de la demande. Faute de transfert après un certain délai, généralement fixé à six mois, l'État où se trouve l'étranger redevient responsable de l'examen de sa demande d'asile. En France, en 2016, près de 26 000 procédures Dublin ont été engagées sur le territoire national, soit une multiplication par cinq du nombre des « dublinés » par rapport à l'année 2014.

dire : en pratique, le système est aujourd'hui à bout de souffle. Dublin fonctionne tant que les flux migratoires ne sont pas trop importants ; mais, en cas de crise migratoire, la difficulté est majeure. D'après l'OFPRA, la France a enregistré 100 412 demandes d'asile en 2017. Signe de l'ampleur de la crise migratoire, ce nombre est en hausse de 17 % par rapport à 2016 et de 90 % par rapport à 2010. L'ensemble des États « Dublin » connaissent des difficultés dans la mise en oeuvre des procédures de réadmission. En 2016, 3 968 transferts ont été effectivement réalisés par l'Allemagne, sur 55 690 procédures engagées, contre 5 244 par la Suède, sur 12 118 procédures, et 61 par l'Italie, sur 14 229 procédures En réalité, plusieurs facteurs expliquent cet échec. Tout d'abord, je pense au manque de solidarité entre les États : le système pèse particulièrement sur un nombre restreint d'États « périphériques » comme la Grèce, l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, ce qui remet évidemment en cause sa soutenabilité. les stratégies d'évitement des États et aux refus de recueil d'empreintes : seuls 23 % des franchissements irréguliers d'une frontière extérieure de l'Union européenne font l'objet d'un prélèvement d'empreintes digitales, ce qui, bien sûr, nuit gravement à l'efficacité de la base de données EURODAC.

En France, le problème s'est récemment trouvé renforcé par l'impossibilité juridique de placer en rétention les étrangers qui doivent être transférés en application du règlement Dublin : c'est bien là le problème ! Des jurisprudences récentes ont remis en cause tout placement en rétention d'étrangers « dublinés », rendant ainsi leur transfert Avons-nous mal anticipé ? Dans tous les cas, il n'y a pas de rétention possible avant la décision de transfert : le Conseil d'État a jugé, en juillet 2017, que le droit français ne prévoyait pas le placement en rétention des étrangers sous procédure Dublin en amont de la décision de transfert, leur rétention étant seulement possible après notification de cette décision. pas non plus de rétention après la décision de transfert. Depuis mars 2017, la CJUE n'autorise le placement en rétention des Dublinés après une décision de transfert que sous conditions uniquement si le droit national de l'État précise, par des dispositions de portée générale, la définition du « risque non négligeable de fuite », qui justifie un placement en rétention. Un arrêt du 27 septembre 2017 de la Cour de cassation en a tiré les conséquences. Il constate que la France n'a pas défini spécifiquement ce « risque non négligeable de fuite » et interdit donc le placement en rétention des « dublinés ». Naturellement, cette situation doit être réglée, car nous ne pouvons pas accepter le dans ces conditions.

Le texte transmis par l'Assemblée nationale prévoit ainsi onze critères alternatifs permettant, sauf circonstance particulière, de caractériser un « risque non négligeable de fuite ». Il simplifie également le régime d'assignation à résidence des « dublinés » et garantit leur droit à l'information. proposition de loi la semaine dernière, entend répondre aux demandes du terrain et combler rapidement ce vide juridique. Je rappelle que les services de l'État sont aujourd'hui démunis face à l'augmentation du nombre de procédures Dublin et face à leur difficile mise en oeuvre.

La commission des lois, qui entend bien ces demandes, juge effectivement urgent de conforter et d'améliorer l'efficacité des procédures Dublin. Elle a ainsi adopté trois amendements.

à faciliter l'organisation des visites domiciliaires pour s'assurer de la présence d'un étranger assigné à résidence, sans avoir recours à la rétention. En outre, la commission des lois a souhaité sécuriser,

Il lui a semblé absolument nécessaire de contrôler la présence sur le territoire d'individus potentiellement dangereux qui, pour certains, ont été condamnés pour des actes de terrorisme.

de la question migratoire : simplifier substantiellement les procédures, assurer des moyens aux politiques d'asile et d'intégration, redoubler nos efforts diplomatiques pour rendre plus efficaces les expulsions et faire enfin aboutir la réforme du régime d'asile européen pour le rationaliser et pour prévoir davantage de solidarité entre les États membres.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le point de départ de ma réflexion est cette phrase du préambule de la Constitution de 1946, elle-même héritée de la Révolution française Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. » Cette phrase nous rappelle que notre tradition républicaine et nos obligations

Lors de l'examen du dernier projet de loi de finances, le Gouvernement a prévu un effort budgétaire en ce sens, comme le rappelait il y a quelques jours encore le Président de la République à Calais.

Dans un contexte marqué également par les surenchères médiatiques, nos collègues députés du groupe Les Constructifs ont choisi d'ouvrir le débat, avant l'examen du futur projet de loi relatif à l'immigration et à l'asile, sur une question très précise

Il est vrai que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à l'origine de cette proposition de loi ne nous obligeait qu'à mieux définir ce risque non négligeable de fuite en fixant des critères objectifs. cependant également insister sur le fait que le texte qui nous est soumis aujourd'hui nous contraint à réfléchir sur un deuxième point : la pertinence d'élargir la possibilité de placer en rétention administrative des « dublinés » avant même que leur soit notifiée la décision de leur transfert. Si l'on réfléchit à droit européen constant, il est clair que les personnes dont la prise en charge relève d'autres États membres doivent faire l'objet d'un transfert vers ces États, ces États, lorsqu'une décision définitive leur ouvre droit à l'asile, ou contraint l'État responsable à organiser leur retour. Cependant, le placement en rétention administrative de demandeurs d'asile sans que l'on soit certain qu'ils feront l'objet d'une procédure de transfert nous conduit à réfléchir à l'importance que nous accordons au principe de dignité humaine. Le débat est comparable à celui qui avait agité le Conseil d'État il y a quelques années et qui mettait aussi face à face le respect de l'ordre public, d'une part, et celui de la dignité de la personne humaine, d'autre part. À l'époque, le Conseil d'État avait jugé qu'il était stérile de vouloir les opposer, dès lors que la dignité était une composante de l'ordre public. C'est également la position de la grande majorité de mon groupe, dont la volonté est non pas de s'opposer à la mise en oeuvre des procédures de transfert prévues par le règlement Dublin mais de s'assurer qu'ici et là le respect de l'ordre public ne soit pas réduit à son interprétation la plus restrictive, qui n'intégrerait pas la notion de dignité humaine.

L'effectivité du droit au recours est aussi un sujet de préoccupation classique au sein de mon groupe. Le débat portera également sur les critères retenus pour établir le risque non négligeable de fuite, dès lors qu'aucune étude d'impact ne permet d'évaluer le nombre de personnes concernées

Nous avons enfin tous à l'esprit qu'il incombe aujourd'hui au Gouvernement de négocier les nouveaux contours du règlement Dublin, même si la tâche s'annonce difficile. Nous sommes favorables à l'élaboration d'un système plus coopératif, où les États membres ne remplissant pas leur devoir d'accueil de demandeurs d'asile devraient verser des compensations financières aux États les plus accueillants. Compte tenu de la pression géographique inégale que subissent certains États de l'Union, il paraît en outre nécessaire de revoir le principe de responsabilité, en introduisant, par exemple, une meilleure prise en compte du critère des liens effectifs entre le demandeur d'asile et l'État membre. En conclusion, je veux réaffirmer notre soutien au Gouvernement dans les négociations qu'il conduit au niveau européen. En revanche, la position de mon groupe sur ce texte est plus partagée, et dépendra grandement du sort réservé aux amendements qui seront défendus par Josiane Costes.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, deux décisions de justice, l'une européenne et l'autre nationale, ont révélé la fragilité juridique des procédures Dublin.

Il s'agit, d'abord, d'un texte technique. Je veux souligner le travail effectué par l'Assemblée nationale, qui est parvenue à une solution équilibrée. Ce texte, en effet, permet de tirer les conséquences des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation, en précisant les critères objectifs au vu desquels doit s'apprécier le risque non négligeable de fuite. Il garantit également l'efficacité de l'action en permettant le placement en rétention

de l'obligation d'information des demandeurs d'asile sur leurs droits et obligations. Au Sénat, la commission des lois a souhaité compléter le dispositif en ajoutant un douzième critère pour caractériser le risque non négligeable de fuite : le refus de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales. Elle propose également de réduire le délai de recours contre une décision de transfert. Enfin, s'agissant des assignations à résidence, elle souhaite, d'une part, faciliter l'organisation de visites domiciliaires pour s'assurer de la présence d'un étranger assigné à résidence et, d'autre part, sécuriser les assignations à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire. Cette proposition de loi a donc été enrichie dans un souci d'équilibre mesuré. Il ne s'agit pas ici de renégocier le règlement Dublin, ni le régime du droit d'asile et encore moins les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, mais ce texte revêt bien une dimension politique, particulièrement à l'approche de

que le phénomène majeur de ce siècle est la crise migratoire, que celle-ci cristallise des désastres humanitaires et des risques sécuritaires, que la moitié des réfugiés arrivés en Europe ces trois dernières années sont le résultat des guerres, sans doute ratées, de l'Occident. Nous conviendrons certainement aussi que l'Europe, y compris la France, faillit en n'accueillant pas dignement des hommes, des femmes et des enfants qu'elle doit protéger, mais qu'elle ne peut

Les images de la jungle de Calais et de Lampedusa ou les agressions de Cologne font le miel des extrêmes, et conduisent aux succès électoraux que l'on connaît,

Au-delà des incantations, des déclarations de principe, voulons-nous doter notre pays de politiques d'éloignement efficaces, des moyens de réguler les flux sur notre territoire pour accueillir dignement celles et ceux qui ont droit à notre protection ? Approuver ce texte, c'est répondre oui. Ces dispositifs de régulation relèvent de la compétence des États membres de l'Union européenne.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, « proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen », tel est le titre trompeur du texte qui nous réunit aujourd'hui. Proposition de loi visant à la banalisation de l'enfermement des étrangers » ou « proposition de loi visant à affaiblir un peu plus le droit d'asile » : voilà des intitulés qui auraient reflété le véritable contenu de ce texte. En effet, les artifices rhétoriques n'y changeront rien, l'objectif de cette proposition de loi, déposée opportunément par les députés Les Constructifs à quelques mois de l'examen du projet de loi sur l'asile et l'immigration, est uniquement d'augmenter le nombre de placements en rétention pour accroître celui des reconduites à la frontière. C'est un retour à une politique du chiffre, donc, et au tout-répressif en matière de politique migratoire. Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, dois-je, en cette circonstance, vous répéter ce que les défenseurs des droits fondamentaux nous rappellent depuis des mois : la gestion répressive des migrations et le non-respect du droit d'asile ne donnent jamais les résultats que l'on prétend en attendre. D'autres parmi vos prédécesseurs, monsieur le ministre Nous opposera-t-on que toutes ces voix, ces presque cinq cents associations, ces avocats, ces magistrats, ces citoyens, dénonçant une politique d'une dureté sans précédent, mentent, probablement sous l'influence de terribles groupuscules d'extrême gauche ? Dérisoire réponse ! Que dira-t-on alors du Défenseur des droits, qui considère que cette proposition de loi constitue un tournant politique déplorable en termes de respect des droits et des libertés fondamentales » ? Encore un gauchiste Le sujet est grave : il s'agit de priver de liberté des demandeurs d'asile juste pour se donner le temps de déterminer l'État européen par lequel ils sont arrivés en premier et où ils ont laissé leurs empreintes. Il s'agit de priver de liberté des demandeurs d'asile contre lesquels aucune mesure d'éloignement n'a été prise. Comme le rappelle la CIMADE, aucune régression de cette ampleur n'avait jamais été envisagée par le législateur. La rétention n'a pas été pensée pour enfermer les gens à titre préventif, pour les avoir sous la main et pour faire le tri entre bons réfugiés et mauvais migrants. Elle devrait uniquement permettre à l'administration- dans un délai raisonnable et dans le respect des droits fondamentaux -d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire. de loi, qui est dans la droite ligne des positions du Gouvernement, vient heurter les principes fondamentaux du droit autant que nos convictions. Les demandeurs d'asile, même placés en procédure Dublin, sont en situation régulière. Et l'on voterait, sans sourciller, la possibilité de les priver de liberté ? S'ériger contre pareille mesure, mes chers collègues, c'est défendre des valeurs, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, défendre la Constitution Humanité et fermeté », tel est le nouveau slogan lancé par le Président Macron et repris à l'envi par les membres du Gouvernement. Sur la fermeté, pas de doute possible, les promesses sont tenues. Quant à l'humanité, on en attend encore des preuves. On n'en trouvera certainement pas dans un texte consacrant la possibilité d'enfermer les familles avec enfants mineurs, placés en procédure Dublin, alors même que la France a été condamnée six fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour cette pratique. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste s'opposera évidemment avec force à cette proposition Ses membres ne cesseront pas de dénoncer, chaque fois que l'occasion leur en sera donnée, une politique migratoire dont ils ont observé les effets dramatiques à Paris, à Calais, à Ouistreham, à Briançon, à Menton et ailleurs. Comme plusieurs personnalités, pourtant proches de M. Macron, l'ont écrit dans une tribune publiée dans le journal, nous ne nous résignons pas à vivre « le journal, nous ne nous résignons pas à vivre « dans un pays où l'on arrache leurs couvertures à des migrants à Calais. Où l'on lacère leurs toiles de tente à Paris. Où l'on peut se perdre, pieds et mains gelés, sur les pentes enneigées de la frontière franco-italienne. Où des circulaires cherchent à organiser le recensement administratif dans les centres d'hébergement d'urgence. » Comment pourrions-nous accepter que « des Érythréens, des Soudanais ou des Syriens, humiliés dans leur pays, torturés en Libye, exploités par des passeurs criminels, terrorisés en Méditerranée et entrés en Europe par la Grèce ou l'Italie [puissent] bientôt être privés de liberté en France ? » La parole est

de réfugiés. J'ai consulté, en préparant cette intervention, des travaux universitaires avançant le chiffre de 64 millions de réfugiés à travers le monde, l'Asie arrivant devant l'Afrique et celle-ci devant l'Europe, dans une approche strictement quantitative. Dans notre pays, le cap des 100 000 demandes d'asile a été franchi en 2017, ce qui a marqué les esprits. Ces mouvements puissants conduisent à s'interroger sur les États-nations, leur souveraineté, comme sur la notion de citoyenneté. Le sujet est donc complexe ; il renvoie à des questions éthiques ou philosophiques perturbantes. Le droit d'asile, nous le savons, est une règle internationale qui est concrétisée dans la convention de Genève et qui bénéficie d'une protection constitutionnelle dans notre pays. Le Sénat sera toujours le défenseur des libertés individuelles, comme des traditions républicaines, pour reprendre une formule utilisée par l'un des orateurs précédents. Ce que nous examinons aujourd'hui, ce n'est pas la réforme du droit français M. le ministre d'État nous annonce pour dans quelques semaines, entre principe d'humanité et principe de réalité. Nous abordons aujourd'hui une première étape, officiellement strictement technique, en examinant

D'une certaine manière, il est même excessif d'évoquer un droit européen de l'asile. La réalité, mes chers collègues, c'est que les traités ne donnent pas compétence à l'Union européenne en matière de droit d'asile. C'est tout le paradoxe ! Ce domaine relève strictement de la souveraineté des États et des législations nationales.

Le règlement Dublin III est, quant à lui, issu des accords de Tampere, de 1999. Notre déception est donc considérable s'agissant du blocage de toute négociation sur ce terrain, avec les problèmes que chacun de vous connaît quant à la position des pays de l'ex-Europe de l'Est, voire de pays traditionnellement proches du nôtre, ne partagent pas tout à fait nos appréciations et, en particulier, ne sont pas prêts à renoncer à leur propre dispositif. La reconnaissance mutuelle des décisions prises en matière de droit d'asile, seule manière de répondre à la problématique des

sur cette dimension européenne, en amont des discussions que nous aurons sur le futur texte. Techniquement, les propositions qui nous sont faites correspondent effectivement aux enjeux. La première réponse apportée dans la proposition de loi consiste

Il s'agit ici de répondre aux préoccupations du Conseil constitutionnel. La troisième réponse, probablement la plus importante, consiste à définir de manière plus objective les critères permettant de penser qu'il peut exister un risque de fuite, de manière à pouvoir de nouveau utiliser le mécanisme de rétention avant de

de décisions de justice, lesquelles ont simplement tiré les conséquences d'insuffisances rédactionnelles de nos dispositions. Il s'agit de compléter ces dernières et non de contredire les décisions de nos plus hautes juridictions.

Rupture, lorsque le 12 décembre dernier, une circulaire remet en cause la tradition et les principes de l'accueil inconditionnel. Rupture, lorsque vous défendez une proposition de loi qui prévoit l'enfermement de demandeurs d'asile dont le code de l'entrée et du séjour encore, ce texte n'exclut pas l'enfermement de mineurs dans les mêmes conditions, et il prévoit que les demandeurs d'asile puissent être enfermés sans avoir de décision d'éloignement.

Mais ce n'est pas possible ! Le système Dublin ne peut plus fonctionner. Le règlement Dublin a été mis en place avec le système de prise d'empreintes EURODAC en raison de l'instauration de la liberté de circulation dans l'espace Schengen. Comme l'a dit le rapporteur, il visait à empêcher une personne de déposer plusieurs demandes d'asile

Nous avons eu un peu plus de 400 000 demandeurs d'asile en 2013, plus de 600 000 en 2014, plus d'1,4 million en 2015 et un peu plus d'1,2 million en 2016. Avec une population d'un demi-milliard d'habitants, l'Union européenne n'arrive pas à faire face à cette

des femmes et des hommes politiques est de construire cette résilience des opinions publiques européennes. Sans cela, l'Europe sera toujours plus faible face à ses voisins.

en donnant la liberté d'installation dans l'Union européenne à toute personne protégée dès lors qu'elle obtient le statut de réfugié et pas simplement après cinq ans

de donner aux préfets des instructions différenciées, pour que, suivant le parcours précédent des « dublinés », ceux-ci puissent rapidement voir leur demande d'asile traitée en France, en particulier lorsqu'ils n'ont pas déposé de demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne. Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, rendre hommage à Angela Merkel, mais en même temps agir comme Viktor Orbán relève d'une duplicité qui pèsera lourdement sur la crédibilité de la France pour refonder l'Union européenne. Nous refusons une refondation de l'Europe qui remettrait en cause les valeurs et les principes qui sont au coeur de la construction européenne depuis ses débuts. Se battre

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, le régime d'asile européen commun repose sur un principe cardinal : un seul État est compétent pour l'examen d'une demande d'asile. Huit critères hiérarchisés permettent de déterminer l'État responsable de l'examen de la demande. Dans la pratique, c'est à partir des prises d'empreintes digitales des demandeurs, enregistrées dans la base de données EURODAC, que fonctionne principalement le régime Dublin. Pour l'année 2016, ce sont près de 26 000 procédures Dublin qui ont été engagées sur le territoire français, soit cinq fois plus plus qu'en 2014. Aujourd'hui nous constatons que le régime Dublin n'est pas efficace. Tout d'abord, au niveau européen, l'application du règlement Dublin rencontre de grandes difficultés en pesant lourdement sur un tout petit nombre d'États- la Grèce, l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie -, dont certains, pour ne pas être déclarés responsables de la demande d'asile, développent des stratégies d'évitement. Ainsi, seuls 23 % des franchissements irréguliers d'une frontière extérieure de l'Union européenne font l'objet d'un prélèvement d'empreintes digitales. l'échelon national, le droit actuel français ne permet pas le placement en rétention des étrangers sous procédure Dublin avant l'obtention d'une autorisation de transfert, conformément à la volonté initiale du législateur, comme l'a rappelé le Conseil d'État, saisi pour avis par la cour administrative d'appel de Douai. Après une décision de transfert, et pour préparer celui-ci, la préfecture peut placer l'étranger sous assignation à résidence ou en rétention. L'article 28 du règlement Dublin III précise les conditions requises pour décider d'une rétention après l'obtention de l'autorisation de transfert : un risque non négligeable de fuite, caractérisé après un examen individuel de la situation et respectant le principe de proportionnalité, étant entendu que d'autres mesures, comme l'assignation à résidence, peuvent être préférées. Mais un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de mars 2017 a considéré que le placement en rétention d'un étranger « dubliné dubliné » ne pouvait être mis en oeuvre par un État que si celui-ci avait défini, par des dispositions de portée générale, les critères établissant le risque non négligeable de fuite. La Cour de cassation a suivi le même raisonnement et jugé que les critères figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autoriser la rétention de droit commun n'étaient pas suffisants, faute de définition explicite du risque non négligeable de fuite. Aujourd'hui, nos préfectures se trouvent privées de moyens. En effet, elles n'ont plus la possibilité de placer en rétention une personne, même si elle a fait l'objet d'une autorisation de transfert. Cette proposition de loi ne vise pas à résoudre l'ensemble de la problématique migratoire. Il ne s'agit pas non plus de débattre de la régulation des flux migratoires. Enfin, ce texte n'a pas pour objet de revoir les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers sur notre sol. de loi vient tirer les conséquences des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation et apporter une réponse en sécurisant juridiquement la possibilité de placement en rétention après la décision de transfert, et en autorisant dans certains cas le placement en rétention avant l'obtention d'une autorisation de transfert. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants-République et Territoires votera en faveur de cette proposition de loi, dont les dispositions sont à la fois pertinentes et justifiées.

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, nécessité fait loi. Plus que jamais, cet aphorisme latin, fondement de notre construction juridique, est illustré aujourd'hui dans la proposition Depuis septembre dernier, cela a été rappelé précédemment, l'autorité administrative ne peut plus placer en rétention un demandeur d'asile dit « dubliné » lorsque son transfert vers le pays de premier enregistrement est demandé. Le cadre juridique d'intervention est donc réduit, et notre vote d'aujourd'hui est d'autant plus important. Si cette proposition de loi ne résout aucun problème lié à la politique migratoire de notre pays, notamment la situation d'afflux massif de demandeurs d'asile et de demandes de titres de séjour auquel nous sommes confrontés, elle permet de traiter le sort des migrants sous statut Dublin. Comme l'a rappelé M. le rapporteur, que je souhaite une fois de plus remercier de son expertise précise de la situation, le règlement Dublin III est une pierre angulaire de la politique européenne d'asile et un gage de respect du cadre de l'espace de libre circulation. Cela a été dit à de nombreuses reprises, nous sommes aujourd'hui confrontés à la nécessité de faire évoluer au niveau européen notre système d'asile. Pour sauvegarder le principe de l'asile des réfugiés politiques, il est indispensable que nous ayons le courage d'assumer un système d'éloignement effectif des ressortissants étrangers dont les démarches pour intégrer notre nation ont échoué et qui n'ont donc plus le droit de se maintenir en France. Mes chers collègues, une politique ferme en matière d'immigration n'est viable que si elle est fondée sur des piliers solides, sans ambiguïté dans leur mise en oeuvre. Si nous voulons vraiment sauvegarder le système d'asile, ce à quoi, sein du groupe Les Républicains, nous sommes profondément attachés, il faut parallèlement avoir un système d'instruction efficace des dossiers de demande, puis un système de renvoi réel, afin de ne pas laisser persister l'espoir suivi de désillusion. Nous restons à cet égard dans l'attente attentive, monsieur le ministre d'État, du projet de loi sur l'asile et l'immigration que vous nous annoncez. Il est en effet nécessaire de changer rapidement de paradigme en la matière. Ainsi, en matière d'immigration régulière, les circulaires Valls de 2012, qui ont permis d'augmenter les régularisations de près de 32 % en quatre ans, sont toujours en application. Par ailleurs, la politique d'intégration elle-même est en souffrance, ne permettant pas de donner les clés nécessaires aux étrangers souhaitant vivre dans notre pays : le contrat d'intégration républicaine, par exemple, mis en place en 2016, est en panne du fait de la baisse du nombre d'heures de formation linguistique. Quant à la politique de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, dont vous nous dites faire une priorité, le budget pour 2018 lui donne à notre sens peu de chances d'être effectivement mise en oeuvre. Nous notons une baisse de 7 % des crédits dédiés à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, lesquels permettront d'effectuer seulement 14 500 éloignements forcés en 2018, alors que 15 161 exactement ont été exécutés en 2014 et 15 485 en 2015. La Cour des comptes l'a relevé sévèrement : l'exécution des mesures d'éloignement est trop faible. Ainsi, en 2016, moins de 18 % des mesures d'éloignement prononcées ont été réellement exécutées, c'est-à-dire que 75 500 personnes se sont maintenues sur le territoire sans en avoir le droit, dont 53 600 déboutés du droit d'asile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les moyens humains les moyens humains sont insuffisants pour assurer les éloignements nécessaires et les centres de rétention administrative sont sous-budgétisés pour assumer la rétention des personnes dont l'avenir n'est pas en France. Malgré cette réalité chiffrée préoccupante, la proposition de loi que nous allons adopter établit la possibilité de rétention dès avant la décision de transfert d'un demandeur d'asile sous procédure Dublin, contrairement au droit commun actuel de la rétention administrative qui impose une décision de transfert. Nous sommes satisfaits que le refus de donner ses empreintes ou leur altération ou leur altération volontaire soient un critère supplémentaire permettant de caractériser le risque de fuite et donc la mise en rétention. Nous nous satisfaisons également que tout élément dissimulé dans la narration du parcours migratoire soit pris en compte dans la décision de possible mise en rétention. Enfin, sans revenir sur l'historique de la disposition, et pour prévenir tout risque de fuite, il est en effet impératif de redéfinir le régime de l'assignation à résidence des personnes faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, bien au-delà de la question des demandeurs asile « dublinés », dont la France connaît aujourd'hui plus que jamais la réalité, ce sujet est préoccupant pour nos concitoyens et pour tout responsable politique. Émigrer de son pays, quelles qu'en soient les raisons, est naturellement toujours une souffrance pour celui qui est contraint de partir. pays d'accueil, doit aussi savoir définir des règles dans le cadre européen pour le système Dublin. Ce dernier repose sur une idée simple : une personne étrangère à l'Union européenne qui demande l'asile dans un État de l'Union n'a pas vocation à le demander ensuite dans un autre pays de l'Union. Pour cette raison, le groupe Les Républicains votera bien entendu la proposition de loi en

Il repose sur le principe qu'un seul État européen est responsable de la demande d'asile d'une personne ressortissante d'un État tiers. Il s'agit d'éviter à la fois que le demandeur d'asile ne sollicite successivement plusieurs pays européens, mais aussi qu'il ne soit renvoyé d'un pays à l'autre sans que sa demande soit jamais examinée. L'État responsable est celui qui a permis l'entrée ou le séjour du demandeur sur le territoire européen. Adopté le 26 juin 2013, le règlement Dublin III s'applique aux vingt-huit pays de l'Union européenne ainsi qu'à l'Islande, à la Norvège, au Liechtenstein et à la Suisse, ces quatre pays faisant partie de l'espace Schengen. Sa mise en oeuvre par les États se fait en deux étapes. Tout d'abord, la détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile : en effet, l'État d'accueil, après étude du parcours migratoire du demandeur, peut estimer que la responsabilité de l'examen de cette demande relève d'un autre État européen. Il sollicite alors cet État, lui demandant de prendre en charge le demandeur. Ensuite, en cas d'accord de l'État sollicité, l'État requérant peut prendre une décision de transfert du demandeur vers cet État. règlement, la France s'efforce d'assurer efficacement ces transferts. Or deux décisions de justice récentes, l'une de la Cour de justice de l'Union européenne, l'autre de la Cour de cassation, ont privé l'autorité administrative de la possibilité de recourir au placement en rétention. Dans un arrêt du 7 mars 2017, la première cour a estimé que le paragraphe 2 de l'article 28 du règlement Dublin autorisant le placement en rétention n'était pas applicable à défaut d'adoption de mesures d'application par les États membres. En effet, cet article précise que le placement en rétention est possible « lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite » de l'intéressé, tandis que l'article 2 définit ce risque comme « l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite » du demandeur. En s'appuyant sur cet arrêt, la Cour de cassation a estimé que, « en l'absence de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur », le placement en rétention était illégal. Les préfectures se trouvent donc démunies pour assurer l'effectivité des transferts. Mes chers collègues, cette proposition de loi tire les conséquences des arrêts précédemment cités. Elle permet de fixer un cadre clair assurant une mise en oeuvre plus efficace de la procédure Dublin. Elle a été enrichie par la commission des lois du Sénat d'ajouts pertinents permettant de lutter plus efficacement contre les refus de prise d'empreintes digitales, de faciliter l'organisation matérielle des visites domiciliaires, d'accélérer les procédures par la réduction de quinze à sept jours du délai de saisine du juge administratif contre une décision de transfert en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention, et de sécuriser les assignations à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.